La séance est reprise. Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, M. Claude Malhuret, président du groupe Les Indépendants-République et Territoires, a demandé de compléter l'ordre du jour réservé à son groupe du mercredi 12 décembre 2018 par un débat portant sur le thème : « Emplois non pourvus en France : quelles réponses ? Quelles actions ? ». Acte est donné de cette demande. groupe La République En Marche, de la proposition de loi visant à la présentation par le Gouvernement d'un rapport au Parlement sur la mise en oeuvre des préconisations relatives aux éventuels risques liés à l'emploi de matériaux issus de la valorisation de pneumatiques usagés dans les terrains de sport synthétiques, et usages similaires, établies par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail le 18 septembre 2018, présentée par Mme Françoise Cartron et plusieurs de ses collègues

le 18 septembre 2018, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, publiait une note d'appui scientifique et technique relative aux risques- éventuels -liés à l'emploi de matériaux issus de la valorisation de pneumatiques usagés dans les terrains de sport synthétiques et d'usages similaires. Ce document est venu établir un point d'étape attendu sur un sujet d'inquiétude. Mais quelle est cette problématique et quelle est sa genèse ? En tant que maire, j'ai parfois été interpellée sur le type de blessures, et leur fréquence, occasionnées sur les terrains synthétiques. Pendant des années, il était donc plutôt question du type de revêtement et de ses conséquences physiologiques pour les sportifs. Il y a un an- aujourd'hui, presque jour pour jour -, une enquête publiée dans le mensuel est est venue mettre en avant la dangerosité potentielle des granules de caoutchouc utilisés. Ces petites billes, que l'on trouve sur un grand nombre de terrains en France, seulement d'en augmenter la durée de vie, mais aussi de rendre possible une activité continue- 365 jours sur 365 -, contrairement aux terrains dits « naturels ». Il existe donc une demande forte, nous le savons toutes et tous ici, quant à la mise en oeuvre de ces structures en France, comme dans bien d'autres pays. Par une question écrite publiée au le 16 novembre 2017, j'ai souhaité interroger Mme la ministre des sports sur l'existence de risques potentiels pour la santé justement liés aux types de matériaux utilisés dans la fabrication de terrains synthétiques.

À cet égard, une réponse gouvernementale à une question écrite de Mme Pascale Boistard, posée en 2013, soulignait déjà des besoins de précision. A-t-on progressé depuis ? Non, hélas ! Les questions restent toujours les mêmes. Nous demandons simplement que le Parlement, et le Sénat en particulier, en tant que maison des collectivités, soit associé aux différentes études qui s'apprêtent à être menées, et qui ne l'avaient pas été jusqu'alors, ou pas suffisamment. Parce que les élus sont directement concernés, j'ai été destinataire de très nombreuses demandes d'information ces derniers mois, de toutes parts : sportifs, parents, associations Cette démarche législative- c'est l'esprit de ce texte -se veut donc collective et constructive. En réponse à ma question, Mme la ministre des sports indiquait, en mars dernier, avoir pris en compte, d'une part, les préoccupations des pratiquants et des communes, principales propriétaires de terrains de grands jeux en France, et, d'autre part, les incertitudes relevées dans le rapport de l'Agence européenne des produits chimiques. C'est pourquoi une saisine de six ministères, en date du 21 février dernier, a demandé à l'ANSES d'analyser les données et les études disponibles sur ce sujet, d'identifier les préoccupations qui pourraient en résulter et de déterminer les besoins complémentaires afin de réaliser une évaluation des risques. Ce travail a donné lieu à la note que j'évoquais, laquelle établit certaines orientations. Tout d'abord, il est écrit que « les expertises scientifiques ne mettent pas en évidence de risques préoccupants pour la santé, en particulier de risque à long terme cancérogène, leucémie ou lymphome

indiquent l'existence de risques potentiels pour l'environnement ». Mais, une nouvelle fois, elle ajoute que « ces données sont insuffisantes pour caractériser les risques éventuels pour l'environnement et les organismes vivants En introduction et en conclusion, l'Agence précise qu'elle a fourni un « appui » et que ce dernier « ne constitue pas une évaluation des risques sanitaires ». sanitaires ». Il « ne vise donc pas à émettre une conclusion de l'Agence sur l'existence ou l'absence de risques, », mais à « hiérarchiser les besoins de connaissance concernant les différentes situations d'exposition ».

le calendrier d'enclenchement des actions visant à préciser certains volets spécifiques afin d'effectuer une évaluation des risques pour la santé humaine humaine ; la position de la France sur la proposition de restreindre la teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les granulats dans un règlement européen concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques chimiques ; la proposition d'éléments méthodologiques en vue de la conduite d'une évaluation des risques environnementaux à réaliser localement, avant toute mise en place de ce type de revêtement. Alors que ces orientations seront discutées avec les six ministères signataires de la demande d'appui- transition écologique, solidarités et santé, économie et finances, travail, agriculture et alimentation, sports

remette au Parlement un rapport dressant l'état d'avancement de chacune des préconisations établies en septembre dernier. Voilà une semaine, lors d'un débat auquel j'ai participé sur le plateau de Public Sénat, plusieurs constats, que je crois unanimes, ont été dressés par des acteurs aux profils pourtant très différents. Premièrement, les élus expriment une inquiétude forte, relayée par les médias, avec parfois des propos alarmistes. Les élus sont en effet responsables de ce qu'ils installent. Étant en première ligne, ils nous disent avoir besoin d'informations claires et fondées. Deuxièmement, tous ont reconnu que cette note de l'ANSES, qui apporte un début de réponse plutôt rassurante, restait insuffisante en l'état, en particulier sur le volet environnemental. les publics concernés et intéressés sont nombreux : pratiquants, clubs, associations sportives- amateurs et professionnels -, familles et enfants, installateurs, personnes chargées de l'entretien, élus, résidents

Les interrogations sur les risques liés à la présence de granulats de pneumatiques usagés dans certains terrains de sport et aires de jeu, relayées par plusieurs médias et associations, s'inscrivent dans ce contexte d'une élévation générale du niveau de sensibilité de la société civile aux problématiques de santé liées à l'environnement. Sans céder aux postures alarmistes ni méconnaître la légitimité des préoccupations ainsi exprimées, il est indispensable de fonder les décisions publiques sur un diagnostic clair et objectif des risques liés à la présence de produits chimiques dans les usages et les pratiques du quotidien. est précisément l'objectif de la présente proposition de loi, déposée par notre collègue Françoise Cartron et les membres du groupe La République En Marche, qui vise à demander la remise d'un rapport au Parlement, avant le 1 janvier 2020, sur les suites données à une récente note relative aux risques liés à l'emploi de granulats de pneumatiques dans les terrains de sport synthétiques et usages similaires. Six ministères ont en effet décidé de saisir conjointement l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, le 21 février 2018, afin d'identifier les connaissances disponibles sur les risques sanitaires et environnementaux liés à ces substances. Menés dans des délais contraints, les travaux de l'Agence ont conduit à la publication, le 18 septembre dernier, d'une note d'appui scientifique et technique qui procède en trois temps. Dans un premier temps, l'ANSES a analysé une cinquantaine d'études et expertises internationales sur les risques liés aux terrains synthétiques, notamment celles réalisées par l'Agence européenne des risques chimiques et par l'Institut néerlandais pour la santé et l'environnement. En matière de santé, l'Agence constate que la majorité de ces études concluent à « un risque négligeable pour la santé » en ne mettant pas en évidence d'augmentation du risque cancérogène associée à la fréquentation ou à la mise en place de terrains de sport synthétiques. En matière d'environnement, l'Agence constate que les données disponibles évoquent « l'existence de risques potentiels pour l'environnement », liés au transfert de substances chimiques les sols, le ruissellement et les systèmes de drainage des eaux de pluie. Les principales substances relarguées et problématiques en termes d'écotoxicité sont le zinc, les phtalates et les phénols. Dans un deuxième temps, l'ANSES indique avoir relevé « des incertitudes et limites méthodologiques » dans certaines publications, en particulier un manque de prise en compte de la variabilité de la composition des terrains synthétiques, ainsi qu'un manque de données concernant les aires de jeu pour enfants et les terrains synthétiques en intérieur. Dans un troisième temps, l'Agence propose donc des axes de recherche prioritaires afin de consolider les données existantes et de compléter les évaluations de risques sur les sujets nécessitant des investigations plus poussées. Lors des auditions, il nous a été indiqué que ces sujets allaient effectivement être intégrés au programme de travail de l'ANSES pour 2019. L'Agence recommande également une évolution de la réglementation REACH afin d'abaisser la teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques, ou HAP, des granulats de pneus, qui constituent des substances particulièrement préoccupantes. La teneur maximale varie actuellement entre 1 000 et 100 milligrammes par kilogramme de mélange, selon l'hydrocarbure considéré, soit un niveau bien supérieur à celui prévu pour les articles destinés au grand public en contact prolongé ou régulier avec la peau : 1 milligramme ou, pour les jouets, 0,5 milligramme. Indépendamment des risques identifiés, il est donc indispensable de faire évoluer rapidement la réglementation en tenant davantage compte des usages, dès lors que, sur un terrain synthétique ou une aire de jeu, le contact direct du corps avec ces granulats peut également être régulier ou prolongé, en particulier pour les enfants. La question va être examinée au cours de l'année 2019 dans le cadre d'un projet de restriction porté au niveau européen par les autorités néerlandaises, en vue de rapprocher les teneurs applicables aux mélanges de celles prévues pour les articles grand public. Sans méconnaître les enjeux socio-économiques de la filière, il me semble important de tendre vers les niveaux les plus protecteurs possible pour les utilisateurs de ces terrains. Enfin, l'ANSES préconise dans cette note l'élaboration d'éléments de méthode pour mener localement des évaluations d'impact avant la création de nouveaux terrains, compte tenu des risques identifiés dès à présent pour l'environnement. Il existe actuellement un grand décalage entre, d'une part, les inquiétudes relayées récemment par les médias et certaines associations et, d'autre part, l'état des connaissances scientifiques. Aujourd'hui, l'absence conjointe de risque majeur identifié pour la santé et de signalement épidémiologique notable ne suggère pas une application stricte du principe de précaution qui conduirait à renoncer complètement à la création de nouvelles installations ou à interdire l'utilisation de terrains existants. Selon les spécificités locales, la sensibilité de la population à ces questions et la volonté des élus, des solutions intermédiaires existent en matière de prévention des risques. Je pense notamment à la région Île-de-France, qui prévoit, après avoir établi un moratoire sur le financement des projets de terrains synthétiques, de rétablir ce soutien en le conditionnant à des critères spécifiques, portant notamment sur la provenance des granulats, sur la conception des terrains pour éviter leur dispersion dans l'environnement et sur la réalisation de mesures régulières portées à la connaissance des utilisateurs du terrain. En s'inspirant de ces pratiques, une collectivité pourrait décider, à l'avenir, d'insérer des clauses guidées par des considérations sanitaires ou environnementales dans les marchés conclus pour la réalisation de terrains ou d'aires de jeu. La définition d'éléments de méthodologie au niveau national et la diffusion de bonnes pratiques pourront utilement éclairer les élus locaux quant aux différentes solutions dont ils disposent. Pour conclure, et sans méconnaître les réticences de la Haute Assemblée à soutenir les demandes de rapport qui se sont exprimées en commission, la présente proposition de loi nous semble utile pour informer le public et aiguillonner les pouvoirs publics, afin que des suites soient effectivement données aux propositions de l'ANSES. Mme la secrétaire d'État pourra sans doute nous apporter des précisions sur ce point. il nous semble judicieux de définir une clause de revoyure sur le sujet, en l'espèce la remise d'un rapport au Parlement d'ici au 1 janvier 2020. Enfin, comme je l'ai indiqué au début la mise en oeuvre des recommandations de l'ANSES doit permettre d'apporter aux élus locaux des éléments de réponse face aux préoccupations exprimées par les citoyens et des outils complémentaires de prévention des risques, s'ils jugent nécessaire de prendre de nouvelles mesures.

La question de l'impact sur la santé d'un environnement dégradé est une préoccupation croissante parmi nos concitoyens.

en conséquence de notre devoir d'évaluer précisément les impacts de ces substances et de prendre, avec responsabilité, les mesures de gestion qui s'imposent. Comme vous le savez, le Gouvernement a porté différentes initiatives en ce sens, certaines étant toutes récentes. La loi prise à l'issue des États généraux de l'alimentation traite ainsi de l'interdiction de l'incorporation du dioxyde de titane dans les produits alimentaires. Elle contient également de nombreuses mesures relatives aux produits phytopharmaceutiques, notamment l'interdiction des pesticides ayant le même mode d'action que les néonicotinoïdes, ces derniers étant déjà interdits en France depuis le 1 septembre 2018. pense également à la séparation des activités de conseil et de vente de produits pesticides, qui réduira la consommation de pesticides en permettant aux agriculteurs d'accéder à un conseil indépendant.

Elles s'inscrivent bien sûr dans le cadre du plan d'action pour une agriculture moins dépendante aux pesticides et du plan de sortie du glyphosate. Il est également prévu un accompagnement fort des professionnels vers de nouvelles pratiques plus vertueuses. Il s'agit bien de les changer en profondeur. Nous portons également au plan national de nombreuses initiatives en faveur de la réduction des risques liés aux expositions aux perturbateurs endocriniens. La deuxième stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens a ainsi été élaborée en lien étroit avec les parties prenantes durant l'année 2018. Elle sera mise en consultation publique d'ici à la fin de l'année. Je veux aussi rappeler les nombreuses initiatives portées dans le cadre européen. La France a été

qu'il s'agisse de la définition des critères européens relatifs aux perturbateurs endocriniens, d'une évolution des agences sanitaires européennes en vue d'une plus grande efficacité,

l'analyse scientifique et technique de l'Agence, restituée le 17 septembre 2018, « les expertises sur les risques liés à l'exposition de sportifs et d'enfants utilisateurs des terrains synthétiques, ainsi que de travailleurs impliqués dans la pose et l'entretien de ces terrains concluent majoritairement à un risque sanitaire négligeable Compte tenu de certaines incertitudes et de lacunes d'information, l'ANSES a néanmoins identifié dans son rapport plusieurs actions permettant d'améliorer l'évaluation des risques. Le Gouvernement a d'ores et déjà pris le parti de suivre les différentes recommandations formulées. Si les rapports existants examinés par l'ANSES sont rassurants, l'Agence relève cependant un manque de données et une grande variabilité de la composition des granulats. Les études en cours menées par l'industrie européenne, et plus encore par l'EPA, l'agence américaine de protection de l'environnement, permettront d'acquérir rapidement de nombreuses données supplémentaires, notamment sur la composition des granulats de pneus ainsi que sur leurs émissions. Les résultats sont attendus au plus tard pour le début de l'année prochaine. Au regard de leur contenu, nous examinerons si des mesures complémentaires doivent être réalisées. La situation doit dès à présent nous inciter à adopter une réglementation plus stricte. stricte. L'évolution est d'ores et déjà engagée dans le cadre du règlement européen REACH. Une restriction a été proposée par nos homologues néerlandais sur les seuils d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, les HAP, présents dans les granulats de pneus utilisés pour les terrains de sport synthétiques. Les autorités françaises appuieront cette proposition au niveau européen, afin de garantir un niveau acceptable d'émission de ces polluants.

pour objectif d'élaborer un guide de bonnes pratiques pour l'évaluation des risques en vue de l'installation des terrains synthétiques, afin d'en limiter les impacts environnementaux. Il s'agit notamment de prévenir la diffusion dans l'environnement des particules de pneumatiques issues de l'usure des terrains, qui peuvent ensuite se répandre dans les sols ou être transportés par les eaux pluviales et avoir des effets négatifs sur les écosystèmes. Ce travail Ce travail sera réalisé avec l'ensemble des acteurs de la filière. Ses conclusions devraient être connues en septembre 2019. Elles permettront d'appuyer les collectivités dans leurs choix d'équipement pour de telles infrastructures.

la mobilisation aux niveaux européen et national. Une telle approche nous guide pour l'ensemble des questions relatives à la question des risques potentiellement induits par les substances chimiques. Si l'avis de l'ANSES offre une première analyse rassurante,

Je vous remercie

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la proposition de loi dont nous débattons ce soir est symbolique du problème posé par le sujet : études après études, enquêtes après enquêtes, les résultats se contredisent.

temps, elle précise que les études montrent toutes, sans exception, des failles méthodologiques importantes. En parallèle, elle omet d'autres études, certainement aussi faillibles, qui se veulent beaucoup plus alarmantes. Je pense notamment aux travaux des universités de Yale, de Géorgie ou encore d'Amsterdam, qui pointent un certain nombre de risques. telle situation n'est pas étonnante, et ce pour deux raisons. Premièrement, on observe une multitude de prestataires en matière de retraitement des pneus usagés, alors même que l'on parle de 23 000 unités par terrain, de 60 mètres par 100. Plus que cette concurrence libre et faussée, c'est l'absence d'un cadre normatif clair sur les caractéristiques des granulats qui suscite nos inquiétudes. En effet, les normes existantes se concentrent presque exclusivement sur les caractéristiques techniques des revêtements, notamment en matière d'amortissement des chocs. La situation est clairement insatisfaisante de ce point de vue, d'autant que, si certaines fédérations régionales ou nationales ont élaboré des guides et donné des consignes de bonnes pratiques, ce n'est pas le cas de toutes. Par ailleurs, la multitude des acteurs concernés et l'absence de normes laissent craindre des traitements de pneus peu respectueux de tous les principes de sécurité.

Deuxièmement, nous sommes face à une multitude de situations, tant les granulats réagissent à toute mutation environnementale. À ce titre, il faut rappeler les études de l'université d'Amsterdam sur l'effet de l'humidité sur les granulats et leur dilution dans l'environnement immédiat. Je peux aussi citer l'étude australienne de 2015 sur les îlots de chaleur créés par l'itinérance des granulats et sur la réaction des billes face à la chaleur, avec une dispersion dans l'air de particules passant par les voies respiratoires. les voies respiratoires. De fait, il n'existe pas une situation environnementale identique d'un terrain à l'autre. C'est d'autant plus problématique que l'on parle non pas d'un type de terrain unique, mais d'un ensemble de terrains de tailles et de systèmes d'aération différents. Celles et ceux qui sont déjà allés dans un en synthétique, lieu très fréquenté par les jeunes, doivent certainement comprendre nos inquiétudes quant aux problèmes respiratoires dans ces environnements clos. C'est d'ailleurs ce que pointe un chercheur de l'université de Géorgie, qui a fait circuler un robot sur les terrains synthétiques pour récupérer les particules pouvant être inhalées. On se l'imagine bien au vu de ces éléments : il est tout à fait envisageable que 23 000 pneus, 120 tonnes de granulats et 190 substances cancérigènes ou toxiques, même en faible quantité, puissent avoir des conséquences néfastes. Or, je tiens à le préciser, plus que la teneur des 190 substances en question, c'est leur accumulation qui interroge. La question sanitaire ne doit pas dissimuler le risque écologique. C'est d'ailleurs, chose étonnante, le seul point sur lequel l'ensemble des études semble s'accorder : les granulats de pneus ne sont pas satisfaisants d'un point de vue environnemental. Sont en cause les îlots de chaleur, qui déstabilisent les écosystèmes alentour, la dilution des granulats dans le sol du fait de l'humidité et leur itinérance. Vous

au liège, à la fibre de coco ou aux modèles hybrides -, elles coûtent cher. Or les collectivités sont déjà en difficulté financière. Pour ne prendre qu'un exemple,

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous sommes aujourd'hui réunis pour examiner une proposition de loi importante sur le fond, mais quelque peu déroutante au regard de la méthode utilisée, puisqu'il s'agit de passer par la loi pour demander au Gouvernement la réalisation d'un rapport sur la mise en oeuvre de préconisations émises par l'ANSES.

proposition de loi pour continuer à travailler sur le sujet. D'ailleurs, dans de récentes conclusions, l'Agence considère que l'exposition à ces surfaces synthétiques présente un risque sanitaire négligeable, tant pour les utilisateurs que pour les spécialistes qui installent et entretiennent ces terrains.

Aussi, par esprit de provocation, pour mettre le Gouvernement et sa majorité devant leurs paradoxes et afin, surtout, d'enrichir le texte, j'ai déposé deux amendements au nom du groupe socialiste et républicain. Mon premier amendement a

Je vous appelle donc, mes chers collègues, à enrichir cette proposition de loi en votant mes amendements. Je le rappelle, il n'y a pas un rapport plus important qu'un autre. Les deux rapports concernent les travaux de l'ANSES. La

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, chers collègues, résumons-nous : la proposition de loi que nous examinons nous invite à débattre de l'opportunité de demander au Gouvernement un rapport qui sera appelé à être remis au Parlement, afin de débattre de ses conclusions au sein des deux assemblées. Bref, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?

D'une part, la composition des terrains de sport synthétiques et des aires de jeu induit des questions de santé publique, mais aussi environnementales, sur lesquelles nous sommes nombreux à attendre des réponses scientifiques, pour mettre fin aux incertitudes, voire aux inquiétudes. D'autre part, la proposition de loi met en lumière des difficultés relatives à la filière de revalorisation des pneus usagés. La note publiée par l'ANSES à la fin de l'été, à la suite d'une saisine de six ministères, porte uniquement sur l'analyse des études existantes et conclut « à un risque peu préoccupant pour la santé, et à des risques potentiels pour l'environnement ». Toutefois, l'ANSES ne donne pas de recommandations provisoires claires. Elle précise que des travaux de recherche supplémentaires pourraient être et sont même nécessaires. En somme, si les études disponibles tendent à nous rassurer sur le plan de la santé, elles mériteraient d'être complétées par un travail de recherche d'envergure. Puisqu'il est question de santé publique, l'initiative doit, me semble-t-il, être portée par les pouvoirs publics.

On peut d'ailleurs s'étonner que les teneurs maximales en hydrocarbures aromatiques polycycliques, les HAP, de ces terrains ne soient pas déjà alignées sur celles des articles de consommation en contact avec la peau, comme les jouets pour enfants. Au-delà de l'inquiétude engendrée par l'absence de données, le sujet intéresse aussi beaucoup les élus locaux. Ainsi, 10 % des terrains sont aujourd'hui synthétiques, une partie d'entre eux étant Certaines collectivités s'interrogent naturellement sur leurs investissements passés ou à venir. Certaines appliquent également le principe de précaution dans l'attente de réponses scientifiques claires. Elles font aussi appel à des matériaux plus coûteux, mais plus sûrs. sûrs. Les conséquences liées à cette incertitude sont donc importantes pour nos collectivités. En réalité, cette proposition de loi concerne plus largement la question de la gestion des pneus usagés, obligatoire depuis 2002, en vertu du régime de responsabilité élargie des producteurs. Les pneumatiques font naturellement l'objet de réglementations pour leur utilisation sur les routes, mais pas pour d'autres usages. Il faut donc d'abord s'interroger sur l'intégration dans cette filière d'un volet dédié à la protection de l'environnement. Ainsi, la recherche devrait être encouragée, pour réduire la production de pneus non biodégradables et difficilement recyclables et encourager la production de pneus recyclés à partir de pneus usés, au-delà du rechapage, ce que nous ne savons pas faire pour l'instant. Ces questions pourraient trouver leur place dans le futur projet de loi d'orientation des mobilités. La réutilisation ne concernant que 16 % des pneus usagés, l'obligation de traitement de ces déchets a conduit les producteurs à chercher d'autres voies de valorisation. Selon les estimations, 90 000 tonnes de pneus usagés sont ainsi transformées en granulats et intégrées à la fabrication de terrains de sport synthétiques Dans une perspective sanitaire, il faudrait faire évoluer la qualification des déchets valorisés, afin qu'ils ne soient plus soumis aux réglementations du produit d'origine, mais à celles du produit de destination.

granulats. Si nous sommes évidemment favorables à de nouvelles études fiables et solides permettant de répondre clairement aux inquiétudes, le véhicule législatif ne nous paraît pas le bon.

En conséquence, souscrivant sur le fond à l'exigence scientifique et à la nécessaire refonte de la filière, mais regrettant le véhicule législatif retenu, le groupe du RDSE s'abstiendra dans sa majorité sur ce texte.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la présente proposition de loi pose deux questions, qu'il convient de bien distinguer. La première porte sur le fond : le recyclage des pneumatiques dans les terrains de sport et les aires de jeu peut-il présenter un danger sanitaire et environnemental ? La seconde est une question procédurale : ce sujet implique-t-il l'intervention du législateur et, en particulier, la demande d'un rapport du Gouvernement au Parlement ? question de fond, celle du danger invoqué. Toutes les données du problème sont dans le rapport de Frédéric Marchand, que je félicite de l'excellence de son travail, d'autant plus qu'il s'agit d'une question d'une extrême technicité.

Les données scientifiques sont insuffisantes. En l'état actuel de nos connaissances, le risque sanitaire serait « négligeable », mais il y aurait des risques « potentiels » pour l'environnement. Cela a très bien été expliqué. La note de l'ANSES du mois de septembre dernier ne constitue pas une étude nouvelle, mais c'est une synthèse des travaux disponibles. De plus, certaines des études compilées seraient méthodologiquement critiquables. Nous devons donc aller plus loin. Il nous faut améliorer nos connaissances scientifiques du sujet. L'enjeu est important pour nos concitoyens, d'une part, et pour les collectivités, Les premiers s'inquiètent à juste titre. Ils sont de plus en plus nombreux à nous demander l'application du principe de précaution. Le sujet concerne non seulement les terrains de sport, qui sont fréquentés par la population, mais également les

Lorsque l'on parle d'infrastructures publiques aussi populaires et symboliques du lien social que les terrains de sport et les aires de jeu, aucun doute n'est permis. Je le disais, alors que nous sommes en plein Congrès des maires, le problème soulevé par la présente proposition de loi est aussi un enjeu majeur pour les collectivités. S'il apparaît qu'il est préférable de remplacer les revêtements utilisés pour les stades et les parcs publics, qui paiera ? Ce sera la commune, comme toujours ! Et la facture risque une fois de plus d'être salée Notre rapporteur a pris l'exemple d'une commune de Wallonie qui a décidé de faire enlever tous les granulats de pneu de son terrain synthétique, ce qui lui coûtera la modique somme de 50 000 euros, et ce sur la base d'éléments scientifiques et techniques dont la fiabilité est sujette à caution. Quand on sait à quel point l'opinion, à l'heure des réseaux sociaux, des et de la récurrence des scandales sanitaires, est prompte à s'emballer quand on mesure à quelle rapidité la panique peut gagner les esprits, on se rend compte de l'urgence du sujet. Sur la base de telles considérations, faut-il abandonner l'usage des granulats de pneus ou seulement modifier leur composition, ou encore continuer de les utiliser, mais seulement en complément de certains autres matériaux ? Faut-il d'ores et déjà, en application du principe de précaution, suspendre leur usage pour la création de nouveaux terrains ou nouvelles aires de jeu ? Nous ne pouvons pas encore répondre à ces questions, qui sont pourtant essentielles. En résumé, sans amélioration de notre connaissance du phénomène et des autres solutions qu'il serait possible de développer pour remplacer les granulats, nous ne pouvons ni agir ni rassurer. Cela me conduit à la seconde question soulevée par le texte : celle de la méthode. Pour faire avancer les choses, doit-on passer par une loi demandant un rapport ? C'est là que nous sommes plus circonspects.

La Haute Assemblée a développé une réticence devenue quasi épidermique à la demande de rapports. À ces considérations générales viennent s'ajouter deux choses d'une part, d'autres études sont en cours à l'échelon international, en Europe et aux États-Unis ; d'autre part, l'ANSES a elle-même confirmé que ce sujet de recherche figurerait dans son programme de travail pour 2019. Dans ces conditions, pourquoi un rapport et une proposition de loi ? Le choix de tels outils parlementaires n'est peut-être pas le plus judicieux. Selon nous, un débat aurait été plus adapté. Il était en effet important que nous nous emparions du sujet. C'est la raison pour laquelle nous remercions le groupe La République En Marche de nous avoir permis de le faire. Si de nouvelles études sur l'emploi des granulats de pneus sont déjà au programme de travail de l'ANSES, nous espérons que le présent débat et la montée des inquiétudes sur ce sujet contribueront à les placer au sommet des priorités de l'Agence. Plus globalement, s'intéresser aux granulats de pneus conduit à s'intéresser à nombre d'autres substances et produits utilisés dans toutes les infrastructures fréquentées par le public : peintures, colorants, colles, agents lissants, Nous sommes en permanence exposés à des substances industrielles dont nous savons finalement peu de chose. Le chantier de la prévention sanitaire est colossal, mais il est vital pour éviter à l'avenir de nouveaux scandales sanitaires de type amiante ou bisphénol. Nous devons nous donner les moyens de le mener à bien. En l'occurrence, puisque c'est surtout l'alerte qui compte et puisque l'adoption d'une proposition de loi ne nous semble pas de nature à faire vraiment avancer les choses, le groupe Union Centriste s'abstiendra sur ce texte. La parole est

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous examinons une proposition de loi visant à demander au Gouvernement un deuxième rapport sur la mise en oeuvre des préconisations d'un premier rapport publié en juin dernier par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Ce dernier visait à clarifier les éventuels risques sanitaires liés à la fréquentation par les sportifs et les enfants des terrains de sport synthétiques et des aires de jeu. En effet, ces terrains, composés de granulats de caoutchouc recyclés à partir de pneus usagés, pourraient se révéler cancérigènes pour l'homme et toxiques pour l'environnement. Cette inquiétude, relayée par les médias, la société civile et un certain nombre d'élus locaux, a conduit le Gouvernement à saisir l'ANSES. Sur la base d'une cinquantaine d'études internationales, cette dernière indique à la fois l'existence d'un risque sanitaire négligeable et la présence de risques potentiels pour l'environnement. Certaines substances chimiques présentes dans ces granulats seraient susceptibles de contaminer les sols et les nappes phréatiques. Néanmoins, elle émet d'importantes réserves d'ordre méthodologique : les données exploitées ne sont pas suffisamment solides pour caractériser la présence ou l'absence de risque pour la santé et pour les écosystèmes. Aussi la portée de ce premier rapport se limite-t-elle à un certain nombre de recommandations, dont la nécessité d'établir des études plus spécifiques et plus poussées. Le second rapport qui fait l'objet de cette proposition de loi permettra, nous l'espérons, d'apporter une réponse claire aux nombreux élus locaux, sportifs et parents d'enfants exposés à ces substances potentiellement nocives pour l'homme et pour l'environnement. Les élus du groupe Les Indépendants sont conscients de l'importance de ce sujet, pour des raisons à la fois sanitaires et environnementales, mais aussi financières. Il ne s'agit pas de faire de la démagogie en demandant aux élus de remplacer demain des terrains dont on vantait hier la qualité et la soutenabilité sans éléments sérieux. Aussi devons-nous clarifier la situation tout en veillant à accompagner financièrement les élus locaux s'il se révélait nécessaire de remplacer ces terrains. Si je soutiens une telle demande de rapport, c'est aussi pour protéger les élus locaux de ce qu'on appelle pudiquement la « faute non intentionnelle

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, les terrains de sport et les aires de jeu dites « synthétiques » sont de plus en plus répandus sur le territoire national. Leur utilisation très pratique pour les clubs et les pratiquants, les économies d'entretien ainsi permises et la valorisation en granulats des déchets de pneus constituent des atouts indéniables. Mais ce type d'équipement suscite également quelques inquiétudes. La proposition de loi déposée par notre collègue Françoise Cartron et le groupe La République En Marche vise à donner une suite à la note de l'ANSES du 18 septembre dernier sur la dangerosité desdits granulats de pneus utilisés pour les terrains de sport. Disons-le tout de suite, l'Agence ne met pas en évidence de risques pour la santé. Elle précise toutefois que son travail « vise à identifier les besoins de connaissance ». Pour lever les doutes, la proposition de loi demande la publication d'un rapport au Parlement qui vérifiera la mise en oeuvre des préconisations du rapport précité de l'ANSES- je souscris parfaitement à la description kafkaïenne qu'a faite notre collègue Nicole Bonnefoy. Ce texte contient deux aspects : un aspect sportif et un aspect relatif au principe de précaution, qu'il soit sanitaire ou environnemental. Sur le plan sportif, l'histoire du gazon synthétique ne date pas d'hier, puisqu'elle est née en 1910 : un chercheur anglais avait fait breveter un tapis tissé de fourrures animales principalement utilisé jusqu'alors pour les décors de théâtre. Dans les années quatre-vingt, l'industrie a commencé à concevoir du gazon synthétique, pour le football en particulier. Les systèmes ont été conçus avec du poil court et un remplissage de sable. C'était pour le moins brutal et traumatique- Christophe Priou a évoqué le sujet. Rassurez-vous, je ne vous imposerai pas la vision des stigmates que porte sur les ischio-jambiers un pratiquant émérite de cette époque que les moins de quarante ans ne peuvent pas connaître Dans les années quatre-vingt-dix, afin de pallier ces effets traumatiques divers, les premiers systèmes de gazon synthétique avec remplissage de caoutchouc ont été introduits. Depuis lors, le confort du joueur et la réduction des divers traumatismes sont devenus de plus en plus importants dans la conception du gazon synthétique. L'Union des associations européennes de football et la Fédération internationale de football association, ainsi que de nombreuses fédérations nationales soutiennent résolument son développement. Par exemple, la Fédération française de football classe et aide au financement d'environ 300 terrains synthétiques par an.

Différents matériaux existent. L'évaluation du risque porte principalement sur les terrains synthétiques qui utilisent un matériau de remplissage en granulats élastomères noirs provenant du recyclage de pneus usagés. De nombreuses études ont été réalisées. Aucune ne conclut à un risque, que ce soit par inhalation, contact ou ingestion. Cela n'exonère pas d'appliquer les principes d'hygiène élémentaire, qu'il faut rappeler et respecter sur tout type de terrain : prendre une douche, douche, se nettoyer les mains et le visage, désinfecter les plaies, se changer complètement après l'entraînement et laver l'équipement utilisé. La dernière étude a été réalisée par, ou ECHA, saisie par la Commission européenne. Les conclusions parues au mois de février 2017 sont claires : il n'y a pas de preuve scientifique d'une augmentation du risque de cancer lié à l'impact des hydrocarbures aromatiques polycycliques, ou HAP, généralement mesurés dans les terrains de sport européens. Le règlement des terrains de la Fédération française de football conseille, en cas de doute et par principe de précaution, ou bien encore dans le cadre d'un suivi sanitaire, de pratiquer des tests. La Fédération continue, en temps qu'utilisatrice de ces surfaces ses clubs affiliés, de s'assurer du respect des normes de construction des terrains en gazon synthétique en vigueur et de s'informer des travaux d'investigations en cours, notamment à l'échelon européen. J'en viens au risque environnemental. Nul ne doute qu'une escouade d'experts dûment accrédités et payés grassement par le contribuable trouvera une de ces fameuses billes dans l'océan.

Je ne peux que constater que nous assistons à une inflation du nombre de rapports promis, lesquels finissent invariablement en classement vertical. Madame la secrétaire d'État, je suis certain que vous aurez à coeur de vous attaquer avec pragmatisme à une telle situation. Mais, de grâce, ne pénalisons pas le développement de la pratique sportive en général et du football en particulier,

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, notre collègue Françoise Cartron a déposé une proposition de loi demande au Gouvernement un rapport sur les risques liés à l'emploi de matériaux issus de la valorisation de pneumatiques usagés dans les terrains de sport synthétiques. 3 millions de pneus arrivent en fin de vie en France, ce qui représente 400 000 tonnes de pneumatiques usagés qui, depuis l'interdiction de mise en décharge par la directive européenne de 1999, sont récupérées par les producteurs de pneumatiques en vue de leur revalorisation. Il en existe trois types : la réutilisation, c'est-à-dire la fabrication de nouveaux pneus, qui concerne environ 20 % des pneus usagés, le combustible, qui en concerne 40 %, et, enfin, la granulation pour la confection de sols sportifs et terrains de jeux pour C'est ce dernier type de valorisation qui pose problème et fait débat. Ces sols et terrains sur lesquels évoluent des sportifs et s'amusent des enfants sont constitués à 90 % de pneus réduits en poudre, mélangés à 10 % de résine. Or, depuis quelques années, une inquiétude est née quant à l'impact sanitaire et environnemental desdits terrains. il n'existe pas de réglementation encadrant la composition chimique de ces granulats. Les normes se concentrent principalement sur les performances techniques attendues durabilité, perméabilité à l'eau, rebond de la balle, absorption des chocs. Le seul test effectué est celui du drainage des métaux lourds. C'est inquiétant quand on sait que certaines des substances chimiques relarguées depuis ces granulats sont des substances nocives, telles que des perturbateurs endocriniens comme le DBP, le DEHP D'autres substances sont utilisées pour accroître les performances des pneus, mais il est presque impossible d'obtenir des informations à leur sujet, étant donné que le secret professionnel protège leur fabrication. À cela s'ajoute le fait que, à côté des granulats, très peu d'études ont été réalisées sur les sous-couches et autres matériaux utilisés dans le processus de fabrication de ces terrains, colorants, les agents liants et lissants, ou les agents anti-UV. Ces terrains sportifs et aires de jeu sont soumis à une utilisation intense et, donc, à une usure mettant en contact direct et prolongé les usagers, en particulier les enfants, Il en va de même pour les pesticides, détergents et autres produits de nettoyage de surface utilisés pour l'entretien des terrains, qui peuvent présenter un risque pour l'environnement et la santé des utilisateurs. Parmi les composants des granulats, on trouve des composés organiques volatils qui, surtout en milieu clos, peuvent provoquer irritations oculaires, respiratoires et cutanées. véritable danger pour la santé publique. Certains producteurs de terrains synthétiques proposent des granulats encapsulés pour limiter la pollution. Il faudrait néanmoins s'assurer que ces capsules ne sont pas responsables d'une pollution supplémentaire s'ajoutant à celle des substances présentes dans les granulats. Ainsi, il demeure des incertitudes sur les risques pour l'environnement et la santé, ainsi qu'un manque de cadre pour évaluer efficacement les risques liés aux composants des pneumatiques. Face à ce risque, six ministères français ont demandé un appui scientifique et technique, en septembre dernier, à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, Cette dernière a analysé les études et expertises actuellement disponibles sur le sujet, fournissant un travail qui ne visait pas à émettre une conclusion sur l'existence ou l'absence de risques. Son rapport insistait bien sur les problèmes méthodologiques de ces études et sur le manque de données. Étant donné que les mesures à prendre relèvent du pouvoir réglementaire et non du pouvoir législatif, il aurait été préférable que ce soit le Gouvernement ...

exact du texte. Pour autant, la question des effets combinés est un vrai sujet qui mérite d'être approfondi. Différents travaux sont en cours aux niveaux national et surtout européen pour mettre en place une méthodologie fiable de mesure de ces effets. Je pense notamment aux projets Euromix et HBM4EU, auxquels participe d'ailleurs l'ANSES. En outre, le Gouvernement s'est déjà formellement engagé à soutenir la recherche dans ce domaine dans le cadre du plan d'action sur les produits phytopharmaceutiques et une agriculture moins dépendante aux pesticides, qui a été publié le 25 avril 2018. Le projet de plan Écophyto II +, présenté aujourd'hui même par le Gouvernement, confirme cet engagement en faveur de la recherche. C'est l'axe 2 du plan en vue de permettre une intégration de ces enjeux lors de l'évaluation des risques préalables aux décisions d'autorisation prévue dans son axe 3.

l'avis du Gouvernement ? Cet amendement vise à étendre la demande de remise d'un rapport du Gouvernement à la mise en oeuvre des préconisations de l'ANSES et à la prise en compte des effets cocktails, en particulier pour les produits phytosanitaires. La prise en compte des effets cocktail est effectivement une préoccupation majeure. Elle constitue un défi

d'un élément fort sur lequel le Gouvernement travaille et s'engage. La question de la prise en compte des effets cocktails est effectivement posée, tout comme la possibilité de mener des études indépendantes pour les dossiers les plus sensibles.

pour répondre à cette question. De même, la France milite pour que les menaces émergentes pour la santé, telles que les effets combinés, figurent en bonne place dans les préoccupations visées par le projet de stratégie européenne pour un environnement non toxique. En France, la question des effets cocktails constitue aussi un enjeu majeur et un vrai défi pour l'ANSES. Afin d'apporter un certain nombre d'éléments de réponse, l'Agence mène le projet PERICLES : financé par l'Agence nationale de la recherche, celui-ci a pour objectif de développer des méthodes pour déterminer les principaux mélanges de pesticides auxquels la population française est réellement exposée son alimentation et d'appréhender les effets combinés potentiels des substances en mélange. Plus largement, l'ensemble de nos organismes de recherche, l'INRA, l'INSERM et l'INERIS, ainsi que de nombreux laboratoires universitaires sont aussi très mobilisés sur cette question. Il s'agit en effet d'un enjeu vaste et complexe, qui nécessite de larges efforts en termes d'investissement scientifique et de travail collaboratif de la part de la communauté scientifique pour contribuer à de possibles évolutions futures de la réglementation. Il s'agit d'un défi scientifique et technique. Pour en revenir à la question de l'usage et de l'incorporation de matières synthétiques dans les terrains de sport, initialement visés par la proposition de loi, il me semble que ce texte a d'abord pour objet d'apporter une réponse pragmatique aux nombreuses inquiétudes exprimées par le public et les collectivités locales. Y associer une thématique relative à la connaissance des effets cocktails relevant encore largement du domaine de la recherche me semble brouiller le message de cette proposition de loi. Cependant,